La séance est reprise. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2020 n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun. Nous reprenons

qui a notamment permis de faciliter la sortie de l'indivision outre-mer, en permettant à une majorité d'indivisaires- vous l'avez rappelé -de procéder à la vente ou au partage de biens indivis pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans. Cet amendement, qui vise à

publics fonciers et d'aménagement de Guyane et de Mayotte soient désormais élus par le conseil d'administration en son sein. Nous n'y sommes pas favorables. En effet, dans tous les établissements publics fonciers ou d'aménagement le ministre chargé de l'urbanisme désigne soit le président, soit au moins un vice-président, ce qui est la moindre des choses. Par conséquent, la commission émet

Cet amendement vise à étendre à Saint-Barthélemy les règles de prescription acquisitive introduites par la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer, qui ramènent à dix ans le délai de contestation des actes de notoriété acquisitive publiés avant le 31 décembre 2027. Initialement, eu égard aux caractéristiques foncières de Saint-Barthélemy, cet article ne lui avait pas été étendu. Mais, à la faveur des règlements successoraux, il apparaît en général qu'il reste des parcelles dont les propriétaires ne disposent pas de titre. Cela s'explique soit parce que les transmissions successives se sont effectuées en passant non pas par un acte notarial, mais par des plans, soit parce que la propriété a tout simplement été établie par la possession.

un dispositif dérogatoire visant à faciliter la sortie du désordre foncier dans plusieurs collectivités ultramarines. En vertu de ce dispositif, un acte de notoriété constatant la possession d'un bien immobilier régulièrement dressé et publié avant le 31 décembre 2027 ne peut être contesté en justice que pendant un que pendant un délai de cinq ans. Cela permet, le cas échéant, aux possesseurs de faire jouer les règles de prescription acquisitive de droit commun prévues par le code civil. Cet amendement vise à étendre le dispositif à Saint-Barthélemy.

j'étais ministre, j'avais attiré l'attention des principaux acteurs politiques martiniquais sur le risque de dissymétrie

En effet, si les dispositions du Ceseda étaient déjà applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, seules ses dispositions relatives au droit d'asile étaient applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Le reste du droit de l'entrée et du séjour des étrangers était régi, dans les trois collectivités du Pacifique, par des ordonnances particulières. Il est donc apparu indispensable, tant pour des raisons pratiques- accessibilité, lisibilité et actualisation -que pour des raisons de fond-

Cet amendement a pour objet de mettre fin à cette discrimination. Les visas à validité territoriale limitée, valables à Mayotte seulement, font de ce petit territoire surpeuplé un lieu d'assignation permanente de dizaines de milliers de personnes.

La création de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy a fait suite à la visite du Président de la République, M. François Hollande, qui avait alors annoncé la création d'une caisse locale. En réalité, la caisse de prévoyance sociale est un bureau de proximité rattaché rattaché à la MSA Poitou. Cette organisation a permis d'offrir enfin à la population un service de proximité pour la gestion de la sécurité sociale. En 2014, mon prédécesseur, Michel Magras, avait déposé une proposition de loi dessinant l'épure d'une caisse autonome répondant de manière équilibrée et prudente à l'aspiration d'une plus grande maîtrise locale des règles en matière de sécurité sociale, tout en ne s'affranchissant pas de la solidarité nationale. Il s'agit donc d'un projet longuement mûri par la collectivité, mais il s'est jusqu'ici heurté à l'opposition en opportunité des gouvernements successifs, faisant faisant de Saint-Barthélemy la seule collectivité ayant un statut de pays et territoire d'outre-mer à ne pas disposer de sa propre caisse de sécurité sociale.

-qui font de la collectivité un acteur du financement de la santé. Or, malgré ce contexte financier favorable, l'hôpital est déficitaire. Sur une île aussi exiguë que Saint-Barthélemy et doublement insulaire, chaque fois qu'une solution peut être apportée localement, elle doit être privilégiée. La crise sanitaire l'a confirmé, s'il en était besoin. La remise d'un rapport au Parlement, objet du présent amendement, vise à dresser un état des lieux de l'organisation du système de santé et de la sécurité sociale afin d'éclairer la représentation nationale sur les enjeux du projet d'organisation différenciée de Saint-Barthélemy. Nous sommes convaincus qu'une organisation différenciée compatible avec la solidarité nationale doit permettre la mise en place d'une gestion optimisée au bénéfice de la population.

En Guyane, entre 90 % et 95 % du foncier appartient à l'État. Or l'une des revendications portées par la crise du printemps 2017 était le transfert de terres de l'État aux collectivités et aux populations autochtones. L'État s'est ainsi engagé à transmettre 250 000 hectares aux collectivités territoriales et 400 000 hectares aux populations autochtones. Trois ans après, la mise en oeuvre de ces deux engagements tarde à se concrétiser.

répertorier les parcelles constituait donc un préalable à toute évolution foncière, qu'il s'agisse de gestion des terres ou de transfert de propriété ». Cet amendement vise à traduire la proposition 36 de ce rapport, en précisant dans le code général des impôts que le cadastre doit couvrir tout le territoire de la Guyane.

? Je dois dire que, par le passé et encore récemment, j'ai eu maille à partir avec l'administration fiscale de Guyane concernant l'évaluation des parcelles forestières exploitées par l'ONF.

Cela me semble tout à fait opportun pour éviter que le défaut de délibération expresse d'une commune ne bloque la procédure. L'article introduit par ailleurs une condition de fond : les communes ne pourraient s'opposer à un projet de cession que si les terrains concernés sont nécessaires à la réalisation d'équipements collectifs, à la construction de logements sociaux ou de services publics. Cette condition de fond me paraît suffisamment large pour ne pas limiter substantiellement le droit des communes elle n'a rien d'aberrant, s'agissant de cessions de biens de l'État à l'un de ses établissements publics. J'ai d'ailleurs cru comprendre que cette condition a été introduite sur l'initiative du Conseil d'État qui s'étonnait que la cession des biens de l'État à un établissement public de l'État soit soumise à l'accord d'une personne tierce, ce qui est tout à fait dérogatoire. L'État consacre des moyens considérables au service de l'aménagement des zones urbaines de Guyane une opération d'intérêt national multisites, ce qui est

entre une autorisation d'urbanisme et la règle d'urbanisme applicable. Il participe à la mise en oeuvre du principe de libre administration des collectivités territoriales. L'amendement prévoit que l'établissement public foncier et d'aménagement de Guyane bénéficie d'un régime d'autorisation moins contraignant pour les projets de construction liés à l'habitat situé dans les périmètres de l'opération d'intérêt national.

vise à créer des plans-guides portant une évaluation globale unique et à dispenser, à titre expérimental et pour une durée de dix ans reconductible, les projets de construction réalisés dans le périmètre de ces plans-guides d'une évaluation environnementale.

à travers un dispositif expérimental sur une période de dix ans, à reconnaître la situation d'urgence à caractère civil que constitue la problématique de l'habitat en Guyane. Ce type de situation, prévu au titre II du code de l'environnement transposant la directive du 27 juin 2011, permet d'exclure du champ de l'évaluation environnementale obligatoire les plans et programmes destinés à contribuer à la résorption de cette urgence à caractère civil.

monsieur le rapporteur,

pour commencer à donner, même si ce n'est pas une finalité, tant s'en faut, un cadre juridique à cette île. Je rappelle que cette île est déserte, inhabitée,

? On a bien compris, dans les propos passionnés de notre collègue Folliot, l'attachement qu'il porte à cet îlot de Clipperton. Pour autant, s'agissant du statut, vous comprendrez bien

nous en remettrons donc à une forme de sagesse, qui puise ses racines dans le texte adopté à l'époque à l'Assemblée nationale, mais nous aimerions avoir l'avis éclairé du Gouvernement. Quel est l'avis du Gouvernement ? Je vais essayer

pour une simple et bonne raison : c'est le ministre des outre-mer qui est administrateur supérieur. Certains de mes prédécesseurs s'y sont intéressés, d'autres non. Pour ma part, il se trouve que cette fonction-là me tient à coeur, parce qu'est en jeu une dimension régalienne d'intégrité de nos eaux territoriales. Vous, qui connaissez bien le dossier, en savez quelque chose. Si, aujourd'hui, un administrateur supérieur voulait faire bouger les lignes, il n'y arriverait pas. Je vous le dis comme je le pense. C'est parce que le ministre que je suis prend cette affaire très au sérieux que nous parvenons à une montée en puissance dans le contrôle de la zone, notamment grâce au plan de relance, en lien avec les armées, particulièrement les forces

que nous n'avions pas les moyens, au-delà du texte qui a été voté à l'Assemblée nationale, d'apporter un regard, une expertise complète sur ce sujet.

un premier pas, dans l'espoir que cet amendement fasse son chemin à l'Assemblée nationale et que, finalement, tout cela se retrouve dans le texte final.

La loi du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer a créé, en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, un congrès des élus départementaux et régionaux, composé, comme son nom l'indique, des conseillers départementaux et régionaux. Ce congrès avait, et a toujours en Guadeloupe, pour objectif de délibérer de toute proposition d'évolution institutionnelle, de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'État vers le département et la région concernés, ainsi que de toute modification de la répartition des compétences entre ces collectivités locales. Les congrès de Guyane et de Martinique ont été supprimés à la suite de la création de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane. Des trois congrès initialement créés, seul subsiste le congrès des élus départementaux et régionaux de Guadeloupe. Il me semble que cette institution gagnerait en légitimité et en expertise si elle associait également, avec voix délibérative, l'ensemble des maires de Guadeloupe. Tel est l'objectif de cet amendement. Intégrer les maires, c'est aussi, à travers eux, intégrer les citoyens et tordre le cou à l'idée selon laquelle les débats sur l'évolution institutionnelle et des compétences sont uniquement l'affaire des élus. J'ajouterai, parce que la confusion est fréquente, que la question de l'évolution institutionnelle ne se résume pas uniquement à la fusion des deux assemblées. C'est justement tout l'intérêt de ce congrès élargi que de débattre des choix les plus pertinents. Je terminerai en vous indiquant que cet amendement a fait l'objet d'échanges avec les présidents du conseil départemental, du conseil régional et de l'Association des maires de Guadeloupe, qui, tous, ont accueilli très favorablement cette proposition. Quel est l'avis de la

d'évoquer notre collègue Théophile. Nous serons donc favorables à son amendement, sous réserve de la suppression de la référence à l'article L. 331-15-6 du code de l'environnement, qui a été abrogé.

explication de vote. Je voterai cet amendement, parce que c'est un amendement de bon sens, qui fait coïncider la loi avec ce qui se fait chez nous. Les maires sont systématiquement invités, mais, c'est vrai, avec voix consultative.

pas simplement de manière verticale, de l'État vers les collectivités. Il peut décider de transferts horizontaux,

Les accords de Guyane de 2017 ont prévu la rétrocession de centaines de milliers d'hectares du foncier de l'État, afin de permettre le développement économique et social de la Guyane. Actuellement, l'État possède 95 % du territoire guyanais et la plupart des communes guyanaises ne disposent pas de suffisamment de foncier pour mettre en oeuvre une véritable politique de logement et de développement. Les engagements de 2017 tardant à se concrétiser, il convient de comprendre les raisons de ce retard et de remédier ainsi au blocage qui pénalise l'essor de la Guyane. En réclamant un tel rapport, le Parlement est dans son rôle de contrôle de l'action du Gouvernement.

transparence, sur la question du foncier en Guyane, dont je n'ignore pas qu'elle a beaucoup occupé les discussions ces dernières semaines sur ce territoire.

La parole est à M. Michel Canévet, pour un rappel au règlement.

Mme Sabine Drexler. Le code général des collectivités territoriales précise que le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles, des classes élémentaires et maternelles d'enseignement public, après avis du représentant de l'État dans le département. Si tel est le cas pour l'ouverture et la création d'écoles, les conseils municipaux ne sont néanmoins pas consultés lorsqu'il s'agit d'une fermeture de classe.

Bien entendu, il est très important, et c'est le cas déjà, notamment dans certaines régions, qu'elles jouent un rôle renforcé en matière de politique universitaire, mais il nous semble que le choix qui a été fait est excessif. La suppression de la carte des formations supérieures et de la recherche, qui constitue le cadre d'implantation et de localisation des établissements et des formations et celui des décisions d'accréditation des diplômes délivrés par les établissements, est assez dangereuse. Outre la suppression du cadre, garant de l'égalité de tous les étudiants sur le territoire, l'article prévoit l'association de toutes les régions pour arrêter les priorités de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur. En fait, les régions sont déjà actuellement associées au titre des représentants des collectivités territoriales.

supérieures et de la recherche, puisque cela remettrait en cause le caractère national de l'accréditation des diplômes. Les universités sont des entités autonomes et, comme telles, elles conduisent une politique de formation et de recherche, elle-même soumise à évaluation indépendante. L'État fixe un certain nombre d'éléments stratégiques, déclinés par les établissements. Si un volet territorial a tout son sens, et c'est d'ailleurs ce que prévoit déjà l'article 16 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche, les régions n'ont pas vocation à s'approprier, en tout ou partie, au détriment ou avec l'accord de l'État, l'ensemble des problématiques de l'enseignement supérieur, de la recherche et des universités. L'enseignement supérieur doit rester une compétence de l'État, afin de garantir la cohérence de la stratégie nationale. Si la Conférence des présidents d'université est favorable à la signature par la région d'un volet territorial, lorsque cela est pertinent, elle est opposée à la signature d'un contrat global. Nous demandons donc la suppression de cet article. Quel est l'avis de

faire. Les auteurs des amendements estiment que l'article que nous avons introduit serait de nature à remettre en cause le caractère national des diplômes et des formations.

régionaux au Cneser, en rendant obligatoire la consultation des conseils régionaux sur la stratégie nationale et en faisant des régions des signataires, et non plus de simples associées, des contrats pluriannuels d'établissement ou de site. Cette dernière modification tend à conforter le contrôle exercé par les régions sur l'offre de formation proposée sur leur territoire

sur la stratégie nationale en la matière, et met en place un mécanisme rendant les régions signataires, et non plus associées, des contrats pluriannuels d'établissement ou de site.

Enfin, bien que les collectivités territoriales soient des partenaires essentiels des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, nous considérons que le contrat de site, dans son ensemble, doit demeurer le support de la relation entre l'État et ses opérateurs, c'est-à-dire les universités, pour garantir la mise en oeuvre des politiques publiques menées par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. La signature de ces contrats par les régions ne nous semble donc pas opportune. La parole est à Mme le rapporteur. Madame

qui n'est pas la nôtre. Le fait que l'État joue pleinement son rôle- vous savez que le concept d'éducation nationale nous est cher et est consubstantiel à la République dans ce pays

des élus régionaux au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce qui est incontestablement une bonne chose, au même titre que la consultation des régions sur la stratégie nationale dans ce domaine. En revanche, cet article prévoit

par le ministre chargé de l'éducation pour une période de trois ans. Or, depuis 2017, la fixation des calendriers est devenue bisannuelle, afin notamment de faciliter la mise en oeuvre de la réforme du second degré. Saisi par le Premier ministre sur le fondement de l'article 37 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a jugé que le caractère triennal des calendriers scolaires relevait du domaine réglementaire. Pourtant, un calendrier scolaire pluriannuel de trois ans serait plus adapté aux activités économiques de montagne notamment, car il permettrait aux professionnels et aux élus de montagne de disposer d'une plus grande prévisibilité. Aussi, cet amendement tend à modifier l'article L. 521-1 du code de l'éducation,

Poncet Monge. Les contrats de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles (CPRDFOP) ont récemment fait l'objet d'une redynamisation et d'une consolidation dans le cadre du lancement du plan d'investissement dans les compétences

qui constituent l'un des niveaux d'intégration de ce plan, ne s'adressent pas au public en phase de transition et de reconversion professionnelle. Le présent amendement vise à garantir les transitions et reconversions professionnelles vers les métiers liés aux enjeux du développement durable.

à renforcer les partenariats entre les collectivités locales et les services déconcentrés de l'éducation nationale. En vue d'engager une dynamique allant dans ce sens, cet amendement déposé sur l'initiative de Jean-Yves Roux vise à ce qu'un bilan annuel soit dressé par le préfet de département,

Toutefois, l'élaboration par le préfet d'un rapport annuel sur les relations entre les services déconcentrés de l'éducation nationale et des collectivités territoriales

soit par le préfet, soit par le président du conseil départemental et que les autres niveaux de collectivités territoriales y sont également associés. Il me semble que le bilan que

Le présent article précise en effet que ces diagnostics devront désormais prendre en compte les besoins en matière d'infrastructures répertoriés et, ainsi, inciter les communes et leurs groupements à se saisir pleinement des enjeux qui s'y attachent dans la définition de leur politique de développement et d'aménagement urbains.

Les départements sont le mieux à même, du fait de leur proximité, de leur parfaite connaissance de leur territoire et des partenaires culturels qui le composent, d'encourager et de renforcer, de fédérer les actions artistiques et culturelles, afin de les rendre encore plus accessibles, en particulier à nos jeunes.

Dans le champ de la solidarité territoriale serait élaboré, tous les six ans, en concertation avec l'ensemble des acteurs locaux, un schéma départemental de la solidarité territoriale définissant un programme d'action destiné à permettre un développement équilibré du territoire et une répartition des équipements de proximité. Compte tenu de son champ, ce schéma se substituerait aux programmes d'aide à l'équipement rural. Pour une meilleure coordination de l'action des collectivités territoriales, et parce que le département est, au titre de sa compétence en matière de solidarité territoriale, le premier interlocuteur du bloc communal, les participations financières aux projets des communes et de leurs groupements devraient être compatibles avec ce schéma de la solidarité territoriale.

Je vois un inconvénient à votre amendement : il tend à subordonner la participation financière de la région aux projets des communes

dépenses réalisées localement sur le réseau transféré à la collectivité, et non une fraction déterminée par l'application de critères de répartition à un volume de dépenses constatées au plan national.

Berthet, est satisfait par la rédaction de l'article 6, celui-ci prévoyant des modalités spécifiques de calcul des compensations financières

Berthet. La période de référence prise en compte dans la détermination de la compensation financière des compétences transférées doit garantir que le niveau moyen de dépenses retenu soit représentatif des charges qui seront réellement supportées par les collectivités bénéficiaires du transfert. Une période de moins de trois ans ne permettrait pas une juste appréciation des dépenses de fonctionnement attachées au transfert de la compétence, en particulier en matière de voirie.

Or les dépenses de l'État ont sensiblement augmenté en matière d'entretien des routes au cours des trois dernières années, plus particulièrement en 2020. Il est donc plus favorable de prendre en compte les seules années 2020 et 2021,

Je découvre les qualités d'ingénieur des Ponts et Chaussées de Mme le rapporteur et je me joins à son avis. La

d'éveiller l'attention de tous sur ce transfert de routes, qui reste volontaire, comme Mme la ministre l'a souligné. On le sait, les routes et les infrastructures qui vont avec

Il fallait que chacun ait bien connaissance de la carte des routes, ce qui a été fait. Il fallait surtout que les métropoles, les départements ou les régions intéressés

par la commission consultative sur l'évaluation des charges du Comité des finances locales, des coûts d'exercice et de gestion des compétences transférées aux collectivités territoriales, au plus tard cinq ans après la promulgation de la loi.

par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges du Comité des finances locales, dans les conditions définies à l'article L. 1211-4-1

vote. Madame la ministre, c'est la deuxième vague de décentralisation des routes nationales. La première a concerné des routes de dimension plus départementale ou régionale que nationale,

de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), c'est-à-dire donner aux collectivités cet argent l'année même de la dépense, encouragera les élus locaux à investir. Six

en année . On peut également rencontrer quelques difficultés en cas de programmes pluriannuels et de séquencement des travaux. Enfin, je pense très sincèrement que la dématérialisation doit permettre aux collectivités de fournir plus facilement les documents et d'accélérer le rythme

j'insiste ! Comme l'a dit Didier Marie, c'est une très bonne initiative, indépendamment de ce qu'en pense Mme la rapporteure. Nous voterons pour cet amendement ; son adoption sera une très bonne chose pour les collectivités concernées.

Madame la ministre, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu'à minuit et demi afin de poursuivre l'examen de ce texte. Il n'y a pas d'observation ?

Le projet de loi prévoit ainsi que les effectifs pris en compte sont les emplois pourvus au 31 décembre de l'année -1, sous réserve qu'ils ne soient pas inférieurs aux effectifs présents un an auparavant. Ces amendements visent à changer l'année de référence pour le contrôle de l'évolution des effectifs transférés. Nous proposons de retenir comme date de référence le 31 décembre 2020, en lieu et place de la mention « un an auparavant », afin de garantir aux collectivités territoriales concernées la prise en compte des effectifs de l'État existant avant l'engagement de l'examen du projet de loi.

entre 2022 et 2024, ce qui empêche de fixer dans la loi une date précise. Si nous supprimions cette souplesse, je crains que nous ne défavorisions

bien construit. Il y est question de la prise en compte du coût des agents de l'État qui ne remplissent que pour partie leur fonction dans des services ou parties de services transférés.

Celle-ci permet de refléter au mieux le coût de recrutement des nouveaux agents en début de carrière, qui assumeront leurs fonctions au sein des collectivités territoriales. Juste et équilibrée, cette méthode a été arrêtée

où la charge est identifiable et ne dépend pas des décisions futures de la collectivité territoriale bénéficiaire du transfert. Enfin, la méthode au « pied de corps » permet de prendre en compte la totalité des composantes de la rémunération des agents et assure, conformément à l'article 72-2 de la Constitution, une compensation financière intégrale, respectueuse du principe du coût historique. Au demeurant, la DGF obéit déjà à des règles complexes et ne peut constituer un vecteur de compensation.

44, cet amendement vise à étendre la disposition prévue aux collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon à l'ensemble des collectivités territoriales, de manière que le nombre total d'agents chargés de cette compétence au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert ne soit pas inférieur à celui qui est constaté le 31 décembre, un an auparavant. En outre, l'amendement tend à changer l'année de référence pour le contrôle de l'évolution des effectifs transférés, en retenant comme date de référence le 31 décembre 2020, en lieu et place de la mention « un an auparavant », afin de garantir aux collectivités territoriales concernées la prise en compte des effectifs de l'État existant avant l'engagement de l'examen du projet de loi.

et le transfert intégral des services de l'État. Il y a là une obligation de résultat et d'efficacité- je ne connais pas un fonctionnaire qui contesterait cet objectif. Chaque agent bénéficie d'un droit d'option lui permet, dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret qui emporte transfert, de choisir entre la conservation de son

peuvent à tout moment demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale ou à être réintégrés dans un emploi de leur corps d'origine. Merci, monsieur

Je pense que le service public, c'est soit le service de l'État, soit le service qui est accompli par les collectivités territoriales. C'est pourquoi je veille toujours à éviter les excès